Notre texte répond en partie à de vraies préoccupations. Il se heurte d'ailleurs aux mêmes obstacles que ceux que vous aviez rencontrés à propos d'un texte relatif au contrôle des écoles hors contrat,

l'alignement des statuts des lois de 1901 et de 1905. Contraindre les associations gestionnaires de cultes à adopter un statut, celui prévu par la loi de 1905, serait inconstitutionnel, nous dit-on. Autrement dit,

de la loi de 1905. L'autre option serait d'imposer aux associations régies par la loi de 1901 les mêmes exigences en matière de gestion et de transparence que celles qui s'appliquent aux associations régies par la loi de 1905. Nous ne demandons pas autre chose.

L'enjeu est simple : il importe de former les imams sur le sol français et de façon adaptée aux valeurs de la République. » C'est la raison pour laquelle nous proposons

les conventions signées entre nos ministres français et les ministres du culte de pays étrangers pour la formation théologique des futurs imams de France et la politique officielle des imams détachés.

un socle de notre vie républicaine. C'est exactement ce que propose Françoise Gatel, en s'inspirant du modèle britannique de conseil consultatif des cultes. Je pense que c'est une excellente initiative, et j'espère que la Haute Assemblée votera

et à toutes partout sur le territoire de la République. C'est aux religions de s'adapter à la République et à l'état de droit, et certainement pas à la République de s'adapter aux pratiques religieuses des uns et des autres. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, déposée par nos collègues Nathalie Goulet et André Reichardt pour faire suite à leur excellent rapport rédigé au nom de la mission d'information sur l'islam en France, la présente proposition de loi aborde un sujet à la fois épineux

très posément, avec conviction, que, au Sénat, ce haut lieu de la démocratie, « gardien des libertés », pour reprendre une expression de notre éminent collègue François Pillet, nous devons pouvoir débattre des sujets qui tourmentent notre société. J'affirme avec conviction et force le respect des centristes pour la laïcité et la liberté de conscience. J'affirme avec conviction que le législateur, vivant au coeur de la société, ne peut ni ne doit éviter, esquiver, taire les réalités, quand celles-ci troublent la société. J'affirme tout aussi posément qu'il ne s'agit nullement de stigmatiser un culte, mais de reconnaître l'importance d'une religion qui compte 6 millions de fidèles dans notre pays, de la respecter et de préserver les musulmans eux-mêmes de l'opprobre qui peut naître de la peur et de la crainte de la diffusion du fanatisme, du repli identitaire. Mes chers collègues, qui peut occulter ou nier ces questions urgentes et complexes que sont la structuration du culte musulman, la transparence des financements, la lutte contre la dérive radicale et la formation des imams ? Il n'est de jour sans débat ou article sur la laïcité et l'exercice du culte dans un cadre républicain. Le ministre de l'intérieur, qui est chargé des cultes, a lui-même déclaré mardi, lors d'un dîner de rupture du jeûne du ramadan, que les enjeux sont trop importants pour que l'État s'en désintéresse. Le texte que nous examinons aujourd'hui répond à deux objectifs principaux : rendre obligatoire l'organisation sous le régime de la loi de 1905 de toute association assurant l'exercice public d'un culte ou la gestion d'un lieu de culte, en supprimant ainsi la possibilité d'opter pour le régime plus souple de la loi du 1 juillet 1901

ayant reçu une formation délivrée par une instance cultuelle à la représentativité reconnue par l'État. Mais cette version initiale du texte se heurtait au cadre juridique très contraignant qui régit cette question et porte atteinte à plusieurs principes constitutionnels majeurs majeurs : la liberté de culte, la liberté d'association, la légalité et la nécessité des délits et des peines. C'est pourquoi, en accord avec les auteurs, j'ai proposé des évolutions, qui ont été approuvées par la commission des lois. Elles sont le fruit d'une navigation délicate et serrée

Ces lois sont de grandes oeuvres législatives, du travail d'orfèvre. Elles ont permis à notre pays de traverser le XX siècle dans un climat de paix sociale et religieuse qui honore encore les auteurs. Toutefois, du haut de ces monuments législatifs, plus d'un siècle nous contemple, et force est de constater que la réalité de ce XXI siècle suscite de nouvelles interrogations. Parlons maintenant du texte. Instaurer l'obligation, pour les associations ayant une activité cultuelle de se soumettre au régime de 1905, constitue une ingérence dans l'organisation d'un culte et se heurte au principe de liberté d'association. Or le Conseil constitutionnel a toujours veillé à ce que les associations puissent se « constituer librement », en application d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. La commission des lois a donc, dans sa sagesse, supprimé toute disposition portant atteinte à ce principe. l'obligation de la formation des ministres du culte reviendrait à réglementer l'accès à la fonction de ministre du culte, mais également la célébration du culte elle-même, qui ne pourrait pas avoir lieu en en l'absence de ministre formé. La désignation par décret en Conseil d'État d'une instance suffisamment représentative de chaque culte reviendrait en outre à ce que l'État détermine lui-même quelles sont les instances représentatives. ces propositions constituerait une immixtion très forte dans l'organisation et la célébration des cultes, en complète contradiction avec le principe selon lequel l'État ne reconnaît aucun culte, et contreviendrait au principe constitutionnel de libre exercice des cultes.

de sorte que cette ingérence de l'État dans le libre exercice des cultes ne trouve pas de justification constitutionnelle. La neutralité de l'État à l'égard des religions est telle que, de façon remarquable, il n'existe pas de définition juridique du culte. S'agit-il d'un flou volontaire, de la part du législateur, pour préserver la liberté de conscience ou d'une identification évidente des cultes existants

entre les citoyens dans l'exercice de leur religion, et plus largement entre les religions, selon qu'un culte disposerait ou non de la capacité à former des ministres du culte sur le territoire français.

rémunérés et recrutés par l'État -intervenant dans les établissements pénitentiaires, les centres hospitaliers et les armées, dans le respect du principe de liberté de culte pour des publics empêchés. Cette disposition reprend le contenu du décret du 3 mai 2017 de Bernard Cazeneuve, alors ministre. Ce décret fait actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, avec une possibilité d'annulation, notamment pour incompétence du pouvoir réglementaire sur le sujet. La commission des lois propose en outre d'instaurer un conseil consultatif des cultes placé auprès du ministre de l'intérieur pour favoriser le dialogue entre les pouvoirs publics et les représentants des cultes.

mais assorties de peines différentes et inférieures, au profit de la création d'une circonstance aggravante pour les délits de provocation à la discrimination ou à la violence à caractère racial, de provocation ou d'apologie du terrorisme, lorsque ces délits sont commis dans le cadre d'une réunion pour la célébration d'un culte. Cette circonstance aggravante se justifie par l'influence qu'exerce un ministre du culte ou tout animateur d'un culte sur les fidèles.

Ces troubles et ces peurs conduisent à une laïcité parfois militante et exacerbée, voire radicale et accusatrice, contraire à l'esprit de la loi de 1905, qui définit une laïcité de neutralité. Le Président de la République lui-même a clairement exprimé sa volonté

un chemin de crête entre liberté et respect de la République, pour retrouver l'esprit initial de la laïcité, celui de la paix religieuse et sociale. Ce chemin, c'est celui de l'exercice de la liberté de culte dans l'espace républicain. La parole

la place de l'islam au sein de la société française, sa place comme culte parmi d'autres cultes en France, soumis aux mêmes principes constitutionnels de laïcité, de liberté d'opinion et de culte, d'égalité devant la loi, mais aussi les défis que des expressions radicales, violentes, dévoyées de l'islam font peser sur notre cohésion nationale. Face à ces défis, le Président

La philosophie de cette réforme est claire ; le Président de la République l'a rappelée au mois de juin 2017. D'une part, chaque Français de confession musulmane a le droit de vivre paisiblement sa foi, comme tous les autres Français, dans le respect du principe de laïcité. Cela signifie que chaque Français, partout en France, est libre de croire ou de ne pas croire, libre de pratiquer un culte ou de n'en suivre aucun. Le Gouvernement n'acceptera jamais que ce principe fondateur soit attaqué, remis en cause ou instrumentalisé. Il le fera respecter sans outrance et sans provocation, mais avec la ferme conviction que la laïcité est constitutive de ce que nous sommes : la France. D'autre part, les Français musulmans ont à mener, avec l'ensemble de la société française et avec l'État, un combat commun essentiel, consistant à faire reculer les idées radicales, en particulier chez les jeunes. Ce constat, vous le faites tous comme moi : si la grande majorité des musulmans français adhèrent pleinement aux idéaux républicains et aspirent à vivre dans la concorde, ils ne sont pas, tant s'en faut, les plus entendus

Nul ne peut nier que leur poids, sur internet, dans certains quartiers, mais aussi dans certains lieux de culte, est excessif. Devant cette prédominance des idées radicales, le Gouvernement et le Président de la République refusent tout fatalisme, car c'est notre rôle de protéger l'ordre public et de préserver la cohésion nationale.

Ces obligations, vous le savez, pèsent aujourd'hui sur les associations qui bénéficient de plus de 153 000 euros de dons ; elles pèseront demain sur toutes les associations

En clair, nous convergeons sur les constats, les interrogations, mais, malheureusement, le calendrier de ces réflexions, comme vous l'avez vous-même relevé, chère Nathalie Goulet, s'avère peu compatible

Dans ces conditions, vous comprendrez que le Gouvernement ne peut être favorable à l'examen de la proposition de loi en l'état, sous quelque forme que ce soit. Il me paraîtrait préférable à cet égard que ce texte soit retiré.

d'être associés aux réflexions en cours. Cela me paraît utile, voire nécessaire ; je ne manquerai pas de le faire valoir dans la suite des discussions avec le Président de la République et le Premier ministre. La parole

l'État-« la France, fille aînée de l'Église » -, et, de l'autre, le projet d'Émile Combes, qui visait à empêcher l'Église de fonctionner selon ses propres règles. La loi de 1905 sauvegarde la liberté de chacun. Son article 1 dispose que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »

Mais quelle est la philosophie de la loi de 1905 et quelles étaient les intentions de ses pères fondateurs ? Au-delà du cadre juridique, il existe, me semble-t-il, une ambition morale de concourir à former des « consciences autonomes ». Ainsi, selon Charles Renouvier, philosophe de la République du XIX siècle, aujourd'hui totalement oublié, « la République n'était pas autre chose que la cité des consciences autonomes »,

est le prolongement et la condition de la liberté individuelle de conscience pour les croyants. Est-il nécessaire de rappeler que, à l'époque de l'élaboration tumultueuse de la loi de 1905, le culte musulman était inexistant en France ? Aujourd'hui, l'islam est la deuxième religion pratiquée sur notre territoire, et ses dérives ne vont pas sans poser problème, au point que les réflexions qui tournent autour de cette religion, y compris, bien évidemment, celles du législateur, tendent à en diminuer les effets collatéraux, voire pervers, tout en essayant de la faire cadrer avec l'esprit républicain. C'est dans cet esprit que nous avons publié

guidait n'était pas de donner à la République la tâche de réformer l'islam- cela dépasserait le cadre de la laïcité -, mais d'inscrire l'avenir de ce culte dans la nation française en sorte qu'il ne dépende plus du monde arabo-musulman- Maroc, Algérie, Turquie, monarchies du Golfe -pour le financement des mosquées et des associations cultuelles, voire culturelles, ainsi que pour la formation des imams. Mais venons-en au texte qui nous est soumis. La proposition de loi du sénateur André Reichardt répond à un double objectif : d'une part, l'unification sous le seul régime des associations cultuelles, tel que défini par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905, de toutes les associations chargées de l'exercice public d'un culte ou de la gestion d'un lieu de culte d'autre part, la création d'une qualification cultuelle des ministres des cultes et l'instauration de l'obligation, pour les associations cultuelles, de ne recruter leurs ministres que parmi les personnes titulaires de cette qualification. La question qui se pose est la suivante : est-il possible d'imposer à une association dont l'objet est l'exercice public du culte de s'organiser sous la forme juridique exclusive de l'association cultuelle

centrée sur la connaissance des lois et règles de notre République, avec comme finalité, disons-le, l'inscription de la pratique religieuse dans le cadre républicain, en particulier celui de la laïcité. Cette qualification serait délivrée par une « instance suffisamment représentative Ce second point contrevient au principe constitutionnel de neutralité, dont découle celui de libre organisation des cultes, puisque, dans cette hypothèse, l'État interviendrait dans la reconnaissance d'une instance cultuelle, ce qui va à l'encontre du principe de séparation des Églises et de l'État. De plus, la fonction de ministre du culte n'a jamais été clairement définie et varie considérablement selon les religions pour ce qui est de la lecture ou de l'interprétation des textes sacrés, mais aussi pour ce qui est des comportements à adopter dans la vie de tous les jours en fonction des prescriptions religieuses. Ainsi, si la séparation de l'Église chrétienne et de l'État est déjà en germe dans les paroles du Christ- « il faut rendre à César ce qui est à César » -, comme le démontre brillamment Marcel Gauchet dans, il en va tout autrement dans l'optique d'une lecture littérale de l'islam, puisque cette religion règle, par la,

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, l'organisation des cultes

Les communautés juives autonomes sont remplacées par un consistoire central et des consistoires départementaux composés de laïcs et de religieux. Portés par cet élan et convaincus que leur modernisation passera par la formation de leurs ministres du culte, les juifs inaugureront en 1830 à Metz une école rabbinique, qui sera transférée en 1859 à Paris,

C'est en effet la version la plus libérale de cette séparation qui a gagné : celle d'Aristide Briand, et non celle du « petit père Combes », adversaire déterminé de la religion. Notre laïcité garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, ce que certains ont, hélas ! parfois tendance à oublier lorsqu'il s'agit de l'islam. Les auteurs de la présente proposition de loi estiment nécessaire de s'ingérer dans le fonctionnement du culte musulman, au motif que la loi de de 1905 aurait été rédigée à une époque où le territoire national ne comptait que peu de musulmans, et que seuls les cultes chrétiens et juif avaient fait l'objet, en amont, d'une adaptation aux lois de la République. C'est aller un peu vite, chers collègues : nos colonies, que je sache, étaient soumises au droit colonial, tiré pour beaucoup des lois républicaines appliquées en métropole, et si leurs habitants n'étaient pas, hélas ! des citoyens français, ils n'en étaient pas moins des sujets de droit, qui ont vu leurs pratiques culturelles et religieuses évoluer, elles aussi. L'islam ne nous est pas si « étranger » que certains le soutiennent Auteure, avec Catherine Troendlé, d'un rapport sur la déradicalisation, je suis consciente des conséquences néfastes des replis identitaires ou du développement des thèses salafistes dans certains quartiers abandonnés par les pouvoirs publics. Ces phénomènes ne touchent pourtant pas l'ensemble des musulmans, qui aspirent à vivre leur foi dans la sérénité. Former les ministres du culte musulman est certes une urgence, mais cela ne nous autorise pas à déroger à nos principes laïques. L'initiative doit venir de l'intérieur du groupe concerné si l'on veut qu'elle ait quelque impact. Les possibilités sont nombreuses, il n'est nul besoin d'imposer un modèle unique. Le cas d'autres religions n'ayant pas de clergé en témoigne. L'impuissance des pouvoirs publics face aux financements opaques, notamment étrangers, des édifices cultuels musulmans interpelle davantage. Ils favorisent le développement d'influences fondamentalistes dans certaines mosquées, ainsi que la prolifération de prêches et discours ultra-rigoristes, inspirés par des lectures non contextualisées des textes scripturaires. C'est cet endoctrinement qui doit retenir notre attention, même si les candidats au djihadisme, finalement, fréquentent très peu les mosquées. Un contrôle de la formation des aumôniers, qui sont rémunérés par l'État, est certes possible

de « contribuer à la réflexion sur les conditions de la formation des cadres religieux et ministres du culte » et de « favoriser le dialogue interreligieux ». Y siégeraient deux sénateurs et Y siégeraient deux sénateurs et deux députés. L'ingérence des pouvoirs publics dans l'exercice des cultes préconisée au travers de la proposition de loi contrevient clairement aux principes posés par la loi de 1905, qui sépare strictement les domaines politique et spirituel. La création d'un tel conseil irait à l'encontre de l'esprit même de la laïcité à la française.

où siègent deux responsables par culte, y compris le culte bouddhiste, et qui se réunit tous les deux à trois mois. Chers collègues, restons dans notre rôle.

Faut-il relancer cette guerre d'un État contre des pratiques religieuses ?

De ce point de vue, faisons très attention à ce que nos débats ne fustigent pas nos concitoyens musulmans, en donnant l'impression que c'est parce que les imams ne sont pas correctement formés

madame Goulet, monsieur Reichardt, que « le ministère du culte relevant de chacun des cultes et, dans la religion musulmane sunnite, relevant même du choix de la communauté des fidèles, l'État ne peut en aucun cas conditionner l'exercice de l'imamat à tel ou tel niveau de formation, ni religieuse ni laïque ».

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi tendant à imposer aux ministres des cultes de justifier d'une formation les qualifiant à l'exercice de ce culte déposée par nos collègues Nathalie Goulet et André Reichardt fait suite à la mission commune d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Cette proposition de loi répond à deux objectifs principaux. Tout d'abord, elle tend à rendre obligatoire l'organisation sous le régime de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État de toute association assurant l'exercice public d'un culte ou la gestion d'un lieu de culte, en supprimant la possibilité d'opter pour le régime plus souple de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association. Ensuite, cette proposition de loi vise à restreindre, sous peine de sanctions pénales, l'exercice de la faculté de célébrer publiquement un culte aux seuls ministres du culte ayant reçu une formation délivrée par une instance cultuelle dont la représentativité serait reconnue par l'État. Elle rend ainsi obligatoire la formation des ministres des cultes, afin de préciser le champ d'application des obligations ainsi posées. de cette proposition de loi a vocation à s'appliquer dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour les cultes ne relevant pas du régime concordataire, c'est-à-dire, en premier lieu, l'islam.

Je tiens à saluer la qualité des travaux du rapporteur, notre collègue Françoise Gatel, qui s'est attachée à dégager des solutions alternatives, tout en répondant à l'intention des auteurs de cette proposition de loi. En premier lieu, la commission a supprimé les dispositions du texte posant des difficultés d'ordre constitutionnel au regard des principes de liberté d'association et de liberté de culte. de culte. Elle a toutefois maintenu l'extension, prévue par le texte, de la réglementation relative à la célébration des cultes aux locaux loués par une association cultuelle, et pas seulement aux locaux dont cette dernière est propriétaire ou qui sont mis à sa disposition. En deuxième lieu, la commission a décidé d'instaurer un conseil consultatif des cultes, placé auprès du ministre chargé des relations avec les cultes et comprenant des parlementaires, afin de favoriser le dialogue entre les pouvoirs publics et les représentants des cultes, ainsi que de contribuer à la réflexion sur l'exercice de la liberté de culte et sur la formation des cadres religieux et des ministres des cultes. En troisième lieu, la commission a décidé d'instituer une formation obligatoire civile et civique, sans dimension religieuse et dans le respect du principe de liberté de culte, pour les aumôniers intervenant dans les établissements pénitentiaires, les centres hospitaliers et les armées. En dernier lieu, la commission a modifié le volet pénal du texte, qui pose une difficulté au regard des principes constitutionnels de nécessité des peines et de légalité des délits et des peines, car il prévoit, pour les infractions qu'il crée, des sanctions différentes de celles qui sont prévues pour des infractions identiques existant déjà. La commission a ainsi prévu la création, pour les délits visés par la proposition de loi et pour des délits connexes, d'une circonstance aggravante s'ils sont commis dans le cadre d'une réunion pour la célébration d'un culte, justifiée par l'influence qu'exerce un ministre du culte ou tout animateur d'un culte sur les fidèles. Sont ainsi concernés les délits de provocation ou d'apologie du terrorisme, ainsi que les délits de provocation à la discrimination, à la haine ou la violence, les délits de diffamation et les délits d'injure en raison de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion. Madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat a la mission fondamentale de garantir nos libertés. Aussi, je souscris pleinement aux modifications apportées par la commission, qui visent à trouver un point d'équilibre entre les libertés, d'une part, et la sécurité, d'autre part.

les auteurs de la présente proposition de loi, nos collègues Nathalie Goulet et André Reichardt, ont choisi de traduire dans ce texte une partie des recommandations qu'ils avaient formulées en 2016, dans le cadre des travaux de la mission sur la place du financement de l'islam en France et ses lieux de culte. Si nous pouvons souligner la qualité des travaux de cette mission pour éclairer nos débats, les membres du groupe du RDSE et moi-même n'approuvons pas le texte qui s'en inspire, que ce soit dans sa version initiale ou dans sa rédaction issue de son examen en commission. En effet, vous le savez, notre groupe est fondamentalement attaché à la loi de 1905 et à ses 44 articles visant à organiser la séparation des églises et de l'État dans notre pays. Les dispositions que vous nous proposez d'adopter aujourd'hui relèvent, pour nous, d'un esprit concordataire que nous ne saurions cautionner. Toute modification de la loi de 1905 risquerait de nous entraîner vers des évolutions inutiles et non maîtrisées. C'était d'ailleurs le cadrage retenu par la mission d'information : « La loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. » Premier écueil, l'exposé des motifs de la proposition de loi initiale vise explicitement l'organisation d'un culte en particulier, à savoir le culte musulman. C'est contraire à l'esprit républicain et à l'esprit de neutralité et de séparation. L'État traite tous les cultes avec la même neutralité et considère tous les citoyens à égalité, qu'ils aient ou non une croyance religieuse, qu'ils la pratiquent ou non. De surcroît, nous devons faire face à une situation paradoxale. Alors qu'une étude de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, réalisée en 2016 démontre le recul de la pratique religieuse en France, une petite minorité s'attache à pratiquer son culte de façon plus dogmatique, voire radicale. Vous vous souvenez sans doute, mes chers collègues, des manifestations et processions à genoux, devant le Sénat, au moment où nous votions la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Les questions relatives à l'organisation des cultes relèvent du ministre de l'intérieur.

qui pratiquent des accommodements déraisonnables pour raisons électorales, tels que les prêts de locaux municipaux et autres financements indirects. La question centrale à laquelle nous renvoie l'examen de ce texte, c'est d'abord celle de l'application pleine et entière des lois de la République et des moyens que, collectivement, nous y consacrons. Si nous sommes opposés à l'esprit de ce texte, il n'en reste pas moins que des problèmes bien réels se posent et que notre pays doit y apporter des réponses concrètes, ce n'est pas la politique concordataire que vous nous proposez qui les résoudra. Elle n'aboutirait qu'à créer davantage de situations discriminantes, d'incompréhensions et de sources de contentieux. Juridiquement, nous ne sommes pas désarmés. Les articles du titre V de la loi de 1905 concernant la police des cultes doivent être appliqués fermement. Je pense aux articles 25, 26, 34, 35 et 36. La loi sanctionne tout citoyen appelant à l'exclusion, au communautarisme, ou encore au meurtre. Plutôt que de choisir l'angle privilégié par les auteurs de la proposition de loi, il aurait été plus acceptable, à mon pour rester conforme à l'esprit républicain, de rappeler la pertinence de ces articles de la loi de 1905, qui contiennent déjà des dispositions d'ordre sécuritaire. je vous donne lecture de deux de ses articles. L'article 35 dispose que « si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. l'article 36, « dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable. » Le texte initial de la proposition de loi a été complètement réécrit en commission. Concernant la formation des ministres des cultes, je vous rappelle que celle-ci existe déjà sous forme de diplômes universitaires, dont le contenu des enseignements dispensés n'est, hélas, ni homogène sur l'ensemble du territoire ni certifié d'un point de vue républicain. Ces formations donnent une caution aux ministres des cultes sans pour autant garantir une réelle appropriation des lois de la République. Dans la pratique, je me demande comment les dispositions de votre texte pourraient s'appliquer aux ministres des cultes autoproclamés, comme il peut en exister, par exemple, dans l'église évangélique. Pour conclure, je voudrais revenir sur la création par l'article 3 d'un conseil consultatif des cultes, placé auprès du ministre en charge des relations avec les représentants des cultes. Une fois de plus, dans la logique de la séparation, les membres du groupe du RDSE estiment qu'il n'appartient pas à l'État de favoriser un tel dialogue : l'oecuménisme revient au religieux. Quant aux structures existantes, telles que l'Observatoire de la laïcité, il pourrait être utile de les renforcer dans leur compétence de lanceurs d'alerte, qu'elles n'assument pas suffisamment, éludant une partie de la réalité, la plus conflictuelle, et se gardant bien de donner des recommandations audacieuses. Elles pourraient réaliser un relevé exhaustif des situations contrevenant à la loi de 1905, en ce qui concerne l'exercice des cultes, le statut des ministres des cultes ou encore dans le domaine des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi à mon tour,

Ses deux objectifs ayant été abondamment rappelés par les orateurs précédents, je n'y reviens pas. Je souhaiterais toutefois préciser qu'elle a été cosignée par plus de cinquante sénateurs et sénatrices des seuls groupes Les Républicains et Union Centriste, que j'ai bien voulu solliciter. Je voudrais Je voudrais tout particulièrement remercier ce dernier groupe, l'Union Centriste, d'avoir bien voulu inscrire dans un de ses créneaux de la semaine dite sénatoriale. Je voudrais également remercier Mme Françoise Gatel, issue de ce même groupe, d'en avoir fait le rapport, tout en m'excusant auprès d'elle de l'importance du travail que cela lui a causé.

le texte que nous examinons aujourd'hui est entièrement vidé de son sens. L'article 1 concernant le recours au régime de l'association cultuelle de la loi de 1905 a été supprimé, de même que l'article 4 relatif à l'obligation de formation des ministres des cultes. S'y substitue un article 3 instituant un conseil consultatif des cultes, placé auprès du ministre en charge des relations avec les représentants des cultes. Il va de soi que cette situation ne saurait me convenir, vous l'aurez compris, non pas par orgueil personnel, étant l'auteur du texte d'origine, mais parce que je pense sincèrement que le Sénat rate ici une occasion de faire réellement oeuvre utile.

Ma préoccupation essentielle concerne la nécessité de rendre obligatoire pour les cadres religieux et les ministres des cultes une formation spécifique leur assurant une connaissance des principes civils et civiques, des rites de leur confession et de la langue française. Mes chers collègues, la raison en est évidente il s'agit bien entendu d'éviter que, faute de formation suffisante, des ministres du culte diffusent des messages contraires à la tolérance et au respect des valeurs républicaines. Au-delà,

Je suis en effet personnellement convaincu que c'est par la formation du plus grand nombre que pourront être endiguées les dérives et les politiques opaques mises au jour dans le rapport de la mission sénatoriale précitée. Pour en avoir parlé abondamment autour de moi, je relève que nombreux sont ceux qui sont du même avis. L'opposition à cette mesure se fonde, non pas sur l'inopportunité de l'objectif visé, mais sur son éventuel caractère inconstitutionnel. À cet égard, je me suis personnellement autorisé à saisir de la question deux éminents constitutionnalistes, dont les études, sous réserve de leur accord, pourraient bien entendu être rendues publiques. Leurs conclusions sont moins radicales que les sentences prononcées ici ou là et que j'ai encore entendues à l'instant. Je me permets ici de m'inspirer des analyses de l'un et l'autre de ces deux juristes concernant tout particulièrement le concept de l'ordre public, sur le fondement duquel des restrictions au libre exercice du culte peuvent être apportées, au sens de l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'une part, et de l'article 1 de la loi de 1905, d'autre part. En l'absence de définition de la notion d'ordre public, il convient de se référer à la décision du Conseil d'État du 28 avril 2004, qui a proposé de retenir, pour l'application de la loi du 9 décembre 1905, une acception large de la notion

Le rapport Stasi de 2003, à l'origine de la loi du 15 mars 2004, qui a encadré, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires, soulignait également que, « aujourd'hui, aujourd'hui, la question n'est plus la liberté de conscience, mais l'ordre public », remis en cause par « les tensions et les affrontements dans les établissements autour de questions religieuses ». Quant à la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, dont l'objet est la prohibition du port du voile intégral par les femmes musulmanes, son fondement dans l'ordre public a même été entendu au sens immatériel des exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans la société française. L'ordre public, mes chers collègues, peut donc s'accorder avec la recherche de l'harmonie, éloignée d'une conception répressive. Partant, une telle définition large de la notion d'ordre public, dans son application au champ religieux, et en particulier à l'islam, est de nature, selon les deux éminents juristes précités, à justifier une conception extensive, sinon instrumentale de celui-ci. Et ils considèrent dès lors que la proposition de loi que, avec d'autres, j'ai déposée intéresse bien l'ordre public, au sens où son objet est d'empêcher la propagation de doctrines religieuses radicales incompatibles avec les lois de la République, de la part d'imams autoproclamés, qui échappent au contrôle de la communauté et qui nourrissent naturellement le terrorisme islamique. S'il s'agit, bien entendu, d'une intrusion dans la libre organisation des religions, cette restriction est on ne peut plus « nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé

comme toujours lorsqu'il s'agit de concilier deux exigences constitutionnelles ou conventionnelles- la liberté religieuse, d'une part, et la sauvegarde de l'ordre public, d'autre part -, il appartiendra au juge,

naturellement compétent, aux termes de l'article 34 de la Constitution, pour « fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques

de trouver un moyen de former les cadres religieux et les ministres des cultes, afin que tous les citoyens puissent exercer leur liberté religieuse dans le respect de nos valeurs républicaines. C'est bien là tout l'objet de ce texte. Les mesures répressives, comme on en voit à longueur de textes, ne suffisant pas, il nous faut un

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, voilà un débat passionnant et animé. Je dois vous avouer que, en écoutant les uns et les autres, j'ai plusieurs fois raturé le texte de mon Plus de cent dix ans après le vote de la loi consacrant la séparation des Églises et de l'État, la question de la laïcité et du lien entre l'État et les religions fait toujours débat.

forte. Après l'intense émotion suscitée par les différents attentats de ces dernières années, il faut distinguer entre deux niveaux de problèmes : d'abord ce qui relève, au sens strict, de la laïcité, par exemple le non-respect de la neutralité d'un service public,

Cela touche les plus fragiles, ceux qui sont en quête de sens après des moments de vie souvent difficiles et qui se laissent endoctriner par toutes sortes de prêcheurs.

Ils nous ont permis, avec ce texte, de débattre sur un sujet essentiel, à savoir la question de la radicalisation. Cela dit, la religion relève de la conscience, et la question posée est la suivante : peut-elle être prêchée par tous ? La République doit être capable, effectivement, de proposer un cadre qui limite les dérives. Cependant, l'État ne peut plus tout contrôler. Il s'agit ici non pas uniquement de légiférer, mais de s'assurer de la capacité de l'État à rendre effective cette loi, sans limiter les libertés de chacun. Je regardais, il y a quelques jours, un film fameux, que j'adore,, du réalisateur François Hanss. C'était une bonne révision avant nos débats

Il faut se rappeler que la loi de 1905 a été pensée dès l'origine comme universelle, s'appliquant à la métropole, mais aussi à l'Algérie, aux croyants de toutes confessions, chrétiens, juifs, musulmans, et,

Notre pays doit, bien sûr, faire face aujourd'hui à certaines menaces : le terrorisme, qu'il ne s'agit pas de nier, la radicalisation d'une forme de l'islam ou l'émergence de nouvelles sectes qui mettent en danger notre République. de répondre à ces menaces sans remettre en cause ce principe de liberté. Mes chers collègues, il faut avoir le courage de la vérité, et Mme la ministre a eu le courage de dire tout à l'heure que nous débattions aujourd'hui

Il ne s'agit surtout pas de considérer que l'islam est incompatible avec les valeurs de la République. Nous devons essayer de comprendre comment le lien peut se forger et se renforcer. Et en arrière-plan, on ne peut pas ignorer qu'il s'agit aussi de s'interroger sur la capacité de la France à assimiler des personnes d'origines culturelles et cultuelles diverses. Voilà pourquoi nous ne pouvons ni imaginer ni tolérer que l'enseignement d'un islam radical soit admis dans notre pays. C'est l'absence de cette limite au quotidien qui met en danger nos jeunes et qui crée le terreau d'une certaine forme d'extrémisme religieux dans notre pays. L'islam de France doit être capable de se structurer, mais ce n'est pas à l'État d'imposer cette structuration. L'État doit se contenter de poser la limite du cadre républicain. La conception de la laïcité française est celle d'une République qui ne se mêle pas de l'organisation interne des religions. L'État ne doit pas aller plus loin que de proposer des formations profanes,

ou plutôt d'une plume vive et souple ? Peut-être les deux ... Notre rôle de parlementaire est de garantir à chacun non seulement la liberté de croire ou non, mais aussi l'exerce de sa croyance.L'État doit ignorer les cultes, tout en permettant le libre exercice des cultes et la pratique religieuse de chacun.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons à la fin de la discussion générale, et bien des choses ont déjà été dites.

le message est clair et intemporel : la science et la connaissance contre l'obscurantisme et l'ignorance ; l'esprit critique et le libre arbitre contre l'endoctrinement et le déterminisme. La réalité, néanmoins, est un peu plus complexe que cela, et cette phrase pose deux problèmes au moins : il n'y a jamais eu en France autant d'écoles qu'aujourd'hui, et, pourtant, le nombre de prisons n'a pas diminué pour autant, loin de là ; délinquance et criminalité des jeunes explosent il n'y a plus seulement que les adultes qui passent à l'acte. L'école et l'enseignement ne font pas tout. La présente proposition de loi tendant à imposer aux ministres des cultes de justifier d'une formation les qualifiant à l'exercice de ces cultes, défendue par mes collègues Nathalie Goulet et André Reichardt, prévoit, aux articles 3 et 4, un contrôle par l'État de la définition de la formation et de la qualification des ministres des Dans le contexte que nous connaissons, l'idée est notamment de remédier au recrutement d'imams étrangers, rémunérés par des pays tiers, véhiculant les thèses d'un islam radical, prêchant en langue étrangère, poussant à la haine et encourageant les pratiques discriminatoires sur notre sol. combattre le phénomène pernicieux des imams autoproclamés. Or ces formations proposées à des radicalisés ne les « déradicaliseront » pas forcément. C'est là Si vous considérez que des imams manquant de qualification pourraient tirer quelque bénéfice de ce type de formation, ayez ceci en tête il existait déjà l'an dernier pas moins de quatorze diplômes universitaires de formation sur le fait religieux et la laïcité, offrant une formation au contexte sociohistorique, au droit et aux institutions de la France, à la gestion d'institutions cultuelles et à une approche universitaire du fait religieux, mais les imams étrangers ne s'y sont inscrits qu'en très petit nombre. C'est là Dans la mesure où elle touche au contenu même de la pratique religieuse, je suis rassurée sur le fait que ladite « qualification cultuelle reconnue », dont devront justifier les ministres des cultes, relèvera non pas du domaine de la loi, mais bien de chaque confession, selon des modalités dont celle-ci sera seule juge. Je suis convaincue en effet que l'État n'a pas vocation à contrôler les instituts de formation théologiques, et encore moins à déterminer le programme de leur enseignement. Ainsi, l'idée de créer une faculté de théologie musulmane au sein de l'université publique, comme il est proposé en application du droit local alsacien-mosellan, ne me paraît pas être une bonne idée. Si le problème des imams étrangers radicaux doit, bien sûr, être réglé, l'on se trompe peut-être de cible ; ou du moins, l'on se trompe d'urgence. En effet, ils ne sont pas le canal principal de la peste islamiste qui ravage le monde et notre pays. Amir Amghar, sociologue spécialiste du salafisme et de l'orthodoxie en islam, explique ainsi que ce n'est plus uniquement dans les mosquées que l'on se radicalise aujourd'hui, mais par des rencontres entre individus par interfaces interposées. Les fidèles sont de plus en plus jeunes et sont en recherche d'informations sur l'islam par d'autres moyens, internet notamment. Là est aussi l'un des chantiers principaux. Le problème de la radicalisation et de la violence des jeunes n'est pas uniquement un problème de jeunes. La vraie question est la suivante : pourquoi notre génération d'adultes rencontre-t-elle plus de mal que celle d'hier à apprendre à l'enfant qui grandit à gérer sa frustration, à maîtriser son agressivité et à découvrir d'autres modes de résolution des conflits que le recours à la violence ? Les bébés du XXI siècle ne naissent pas plus violents que ceux des siècles précédents. Le problème central est celui de l'éducation, qui est l'apanage des parents. La formation, l'instruction, si elles peuvent aider à l'insertion dans la société par une accumulation de compétences, ne remplaceront jamais la transmission donnée par le cadre familial, qui, seule, peut marquer durablement un individu et en faire quelqu'un de bon et d'impliqué pour le bien commun. La formation des imams est utile, certes, mais il ne faudrait pas surestimer ses effets. Il convient de garder à l'esprit qu'elle ne constitue pas uniquement la solution ultime au mal du siècle.

En effet, il vise à compléter la seconde phrase de l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Celle-ci indique : « La République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public ».

effet, la notion d'ordre public, dans son application au champ religieux, n'a jamais été définie avec précision, ni dans la loi de 1905, ni dans les discussions parlementaires. Malgré

le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité publique ? Ou faut-il l'entendre aussi au sens immatériel des exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans la société française ?

déjà dans le texte, puisque c'est la liberté du culte et le respect des cultes qui nous mènent au vivre ensemble. Je ne sais pas pourquoi vous vous ingéniez à

elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions éditées, ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. » Votre amendement, dépourvu de toute portée

dans le respect de l'ordre public et de notre Constitution, parce qu'ils y croient et qu'ils croient aussi, comme nous, à la laïcité et à la République ! La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

raisons pour lesquelles je m'interroge sur la première phrase de l'objet de votre amendement : « La laïcité, c'est la liberté, mais c'est aussi l'égalité, l'égalité entre les citoyens quelle que soit leur croyance. »

ici au Sénat, dans le cadre de la loi « Égalité et citoyenneté », pour aligner les obligations comptables des statuts des lois de 1901 et 1905.

si je l'avais dit, cela supposerait que j'aurais osé inviter quelqu'un à entreprendre l'escalade de la loi de 1901 et à redescendre sans parachute, ce qui m'étonne fort

sous réserve d'une dissociation entre les activités strictement cultuelles assurées par une association à objet cultuel et les autres activités exercées par une association généraliste, Nous avons bien compris qu'il n'était pas possible de placer toutes les associations gérant un lieu de culte sous le régime des associations de la loi de 1905. C'est la raison pour laquelle la proposition faite par Mme Goulet vise simplement

! En effet, nous proposons régulièrement que le contrôle du respect de la distinction intervienne aussi au moment de la création d'écoles privées hors contrat, qui sont souvent adossées financièrement à des associations cultuelles de fait,

Le scrutin est ouvert.

Si l'on se réfère à son arrêt du 19 juillet 2011, le Conseil d'État a considéré qu'il était possible à une commune de mettre un local à la disposition d'un culte dans les conditions financières de droit commun, comme pour toute association, et dans des conditions d'égalité de traitement, mais qu'il n'était pas possible de mettre à disposition, de façon pérenne et exclusive, ce local,

de l'amendement, à savoir interdire aux personnes publiques de louer des locaux à une association cultuelle, contrevient à deux libertés fondamentales : la liberté de réunion et la liberté de culte. En dernier lieu, la crainte, exprimée par Mme Laborde, de l'application de tarifs différenciés selon les cultes n'est pas fondée. En effet, pour toute mise à disposition de locaux communaux au profit d'associations, qui en font la demande en application de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, la jurisprudence constante du Conseil d'État interdit que tout avantage soit octroyé à un culte par rapport à un autre, en vertu des principes

qu'il n'y ait pas plus de transparence quant aux obligations statutaires des associations cultuelles : cela n'a rien de stigmatisant et c'est complètement logique. Voilà en tout cas une illustration de la confusion des genres que nous entretenons.

laïque : son régime juridique est celui d'une stricte séparation entre l'État et les cultes. Cette séparation est consacrée par l'article 2 de la loi de 1905, qui a acquis une valeur constitutionnelle. Il découle de ces règles constitutionnelles plusieurs exigences : d'abord, le principe de non-reconnaissance, en vertu duquel aucun culte ne saurait disposer d'un statut de droit public, ni occuper une place dans le fonctionnement de nos institutions. Ensuite, du principe de laïcité, ainsi que du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, découle le principe de neutralité de l'État : celui-ci ne saurait privilégier ou défavoriser un ou plusieurs cultes. Enfin, le principe de laïcité garantit la liberté de conscience. Les pouvoirs publics sont ainsi garants de la liberté du culte, de la liberté d'exercice des cultes, et de leur libre administration. La création d'un conseil consultatif des cultes porterait atteinte à l'ensemble de ces principes. C'est pourquoi

la Grande-Bretagne, où il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Ce modèle communautariste ne me plaît pas, madame Gatel, et je vais vous expliquer pourquoi. Il existe aujourd'hui une religion, le pastafarisme,

auquel je voue un culte particulier ! Quelle sera la position de notre docte Assemblée ou du Conseil d'État, quand, demain, une religion druidique demandera, tout naturellement, à être associée à ce conseil ? Je pense sincèrement que nous entrons là dans des discussions infinies, et qu'il vaut mieux en rester à la sagesse de 1905 : la neutralité absolue nous évite d'ailleurs de définir

Je vous livre ma réelle conviction, avec beaucoup de sincérité et de franchise. Je rappelle qu'il s'agit ici d'un conseil consultatif. Quand le Président de la République, quel qu'il soit,

tout ! Je voudrais en revanche revenir sur la formation des imams. C'est une nécessité- tout le monde le reconnaît, il n'y a pas là de problème -, mais je suggérerai

de l'article 3 . En effet, nous considérons que la création d'un conseil consultatif des cultes porterait atteinte au principe de non-reconnaissance des cultes et au principe de neutralité de l'État, ainsi qu'à la liberté d'exercice des cultes et à leur libre administration, comme je l'ai dit tout à l'heure.

a pour mission de favoriser le dialogue interreligieux. Une telle mission ne peut être conforme au principe de neutralité de l'État, qui interdit à celui-ci, et donc à un conseil placé auprès de lui, de s'immiscer dans la doctrine des cultes, dans leur organisation et dans les relations qui

financés par des pays étrangers sous la forme de détachements de fonctionnaires dans le cadre d'accords bilatéraux. Au passage, bravo pour la laïcité, dont on nous parle depuis par des États étrangers, dont 151 provenant de Turquie, 120 d'Algérie et 30 du Maroc. Rappelons que, par ailleurs, il y aurait au minimum entre 2 500 et 3 000 mosquées dans notre pays. Tous les autres imams sont choisis par la communauté

cette situation n'est pas acceptable et, même si l'islam sunnite, majoritaire en France, est une religion du sacerdoce universel, où chaque où chaque fidèle est un ministre du culte en puissance, ce caractère universel du sacerdoce ne doit pas remettre en question l'importance qu'il y a à disposer d'un encadrement formé, qui maîtrise à la fois la théologie musulmane et le contexte français, et qui soit en mesure de développer un contre-discours face aux discours de surenchère radicale. Précisément parce que tout fidèle peut devenir imam, il faut que la formation des imams puisse faire émerger des cadres qui maîtrisent le texte et s'investissent dans son interprétation, adaptée au contexte français.

Cette qualification et cette formation seraient définies par la confession concernée, après consultation du conseil consultatif des cultes, et non plus par une instance insuffisamment représentative, définie par décret en Conseil d'État.

Si l'État dispose de la faculté d'exercer ses pouvoirs de police administrative dans le but de prévenir les troubles à l'ordre public, ces derniers doivent être suffisamment graves pour justifier d'une telle immixtion dans

Comme je l'ai déjà indiqué, ces conditions sont loin d'être réunies : il faudrait que l'obligation de formation corresponde juridiquement à une exigence d'ordre public. Très sincèrement, mon cher collègue, les obligations

cet amendement pourrait être contesté.

les vrais cadres d'une mosquée ! Ce n'est certes pas à nous d'élaborer le programme de l'enseignement théologique, mais il ne faut pas oublier que les prêches de ces imams pèchent, si je puis

Je relis ce qu'a écrit l'un d'eux : « Il est extrêmement délicat d'anticiper une quelconque réponse, tant de la part du Conseil constitutionnel que de la Cour européenne des droits de l'homme, dans un sens ou dans l'autre Pour ma part, compte tenu des enjeux pour notre pays, je pense qu'il faut prendre ce risque. Le juge constitutionnel ou conventionnel appréciera ensuite, selon la règle dite « du contrôle de proportionnalité ». Certes, une telle mesure implique du courage politique, car il faudra l'assumer,

que nous portons. Si ces personnes avaient revendiqué leurs actes au nom de la religion, nous n'aurions pas épuisé la question de la justification de ces morts.

ma famille ont payé de leur vie, de leur sang, la défense de nos libertés. Je serais prêt à les défendre avec la même vigueur, mais aussi avec les outils de la République. Ceux de la religion ne m'intéressent pas Nathalie Goulet, pour explication de vote. on retrouvera ses dirigeants dans la rue en train d'exiger des lois de plus en plus répressives, des mesures de plus en plus fantaisistes contre les fichés S, des dispositifs totalement extra-juridiques et sans base légale

fallait que la loi républicaine soit appliquée partout et que c'était aux religions de s'adapter à la République, non à la République de s'adapter aux religions. Je partage donc complètement votre position sur les outils républicains, dont vous assurez la promotion à juste titre. Je tiens simplement à dire que la demande d'une formation

4 qui traite des aumôniers et de leur formation. J'ose espérer que les aumôniers embauchés,

et nouvellement recrutés à compter du 1 octobre 2017, d'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée a été instaurée

dans les cultes. Quand certains ont parlé de formation et que j'ai rejeté cette idée, il m'a semblé que nous partagions la même vision des choses.

Nathalie Goulet, pour explication de vote. Je soutiens absolument la position de la commission. Pour avoir présidé la première commission d'enquête sur les réseaux djihadistes, en 2014, dans cette maison, pour avoir visité les lieux privatifs de liberté et avoir rencontré l'ensemble des aumôniers qui y travaillent,

S'il faut reconnaître que l'unification du régime juridique applicable aux associations cultuelles pourrait être justifiée par la volonté de tracer des lignes de démarcation plus claires entre les activités cultuelles et les activités non cultuelles, il serait à mon avis hâtif d'adopter un texte dont l'ossature contrevient manifestement à des libertés de nature constitutionnelle et conventionnelle. Même si une solution de repli plutôt adroite a été trouvée par notre rapporteur, dont je salue le travail, pour instituer une obligation de formation pour les aumôniers intervenant dans les services publics pénitentiaires, hospitaliers et militaires, il n'est pas certain, comme l'a rappelé notre collègue Jacques Bigot, qu'elle relève de l'action du législateur. Je me pose par ailleurs la question de l'opportunité et de la pertinence de ce texte pour les collectivités ultramarines. À Mayotte, mais également en Guyane, la loi de 1905 n'est pas appliquée. En conséquence, proposition de loi avait été adoptée dans sa version initiale, on aurait interdit aux cultes de s'organiser en loi 1901 sans leur permettre de s'organiser en loi 1905. 1905. Seul aurait été possible l'exercice des cultes et des missions religieuses des décrets-lois Mandel, ce qui est une formule peu utilisée. J'attire solennellement l'attention de notre assemblée

non pas la deuxième religion, mais la première religion. Je déplore donc que les auteurs de ce texte n'y aient pas songé, alors que, dans mon territoire, jamais la pratique de l'islam n'a posé de problème vis-à-vis des règles de la République. C'est la raison pour laquelle je voterai contre ce texte.

Le scrutin est ouvert.

tous immeubles », en faisant un bail commercial pour le commerce et un bail locatif à usage d'habitation pour les autres logements, d'interdire la condamnation des issues aux étages et d'appliquer une taxe sur les logements vacants, avec des taux renforcés

du propriétaire, par exemple du fait de l'insuffisance de la demande locale. Cet article nous permettra de remettre sur le marché de nombreux logements aujourd'hui stérilisés au-dessus des commerces. Il ne coûte rien

qui vise à augmenter de 66 % à 75 % la réduction d'impôt sur le revenu pour des particuliers qui mettraient à la disposition d'associations culturelles des locaux à titre gratuit, a fait l'objet d'un avis de sagesse de la commission des finances.

Le plafond de dépenses est identique : 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple, avec des majorations pour personnes à charge. Le crédit est de 15 % des dépenses engagées, contre 15 % à 30 % pour le CITE en fonction du type de travaux.

qui n'en avaient pas forcément le plus besoin, car il était d'autant plus élevé que le bien était onéreux, et contribuait à la hausse des prix, puisqu'il était ouvert à tous les acheteurs. On observerait probablement les mêmes effets avec le dispositif proposé, puisqu'il suit les mêmes modalités. Enfin, et surtout, ce crédit d'impôt a été remplacé,

finances rappelle que les organismes HLM, de même que les autres organismes de logement social, sont déjà exonérés du paiement de l'impôt sur les sociétés pour les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général.

d'exonérer de taxe de publicité foncière et de droits de mutation les acquisitions d'immeubles situés dans les périmètres OSER. Il est rappelé que l'article 1594-0 G du code général des impôts exonère certaines opérations de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement. C'est le cas lorsque l'acquéreur s'engage à reconstruire l'immeuble, ou dans le cadre de zones à urbaniser par priorité ou de zones d'aménagement différé. Tel est le dispositif existant. L'exonération proposée par l'amendement serait beaucoup plus large, puisqu'elle concernerait l'ensemble du périmètre des centres-villes OSER, soit au moins 4 % de la surface urbanisée et une proportion sans doute nettement plus élevée des immeubles. Les droits de mutation sont un impôt certainement critiquable, qui a d'ailleurs été encore récemment l'objet de critiques. Ils ont sans doute un impact social, car ils rendent coûteuse la cession d'immeuble, donc le déménagement pour un propriétaire. Pour autant, leur réforme éventuelle ne peut être faite à l'occasion de cette proposition de loi et devrait intervenir dans un projet de loi de finances, dans le cadre de la réforme des finances locales annoncée par le Gouvernement. Accessoirement, ce serait aussi une perte de recettes importante, non seulement pour la commune, mais aussi pour son département. En conséquence, l'avis de la commission des finances

Les bailleurs sociaux bénéficient d'ores et déjà d'un dispositif fiscal dérogatoire, dans la mesure où les bénéfices se rapportant aux activités réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés d'impôt sur les sociétés. Au regard de la réglementation européenne, ces exonérations constituent une compensation de service d'intérêt économique général exemptée de notification, car elles relèvent de la décision de la Commission du 20 décembre 2011. Les compensations de service d'intérêt économique général sont exemptées de notification, car elles sont présumées compatibles avec le marché intérieur, dès lors qu'elles remplissent les trois critères suivants : l'existence d'un mandat d'exécution des obligations, les paramètres de calcul de la compensation établis préalablement et l'absence de surcompensation. Or rien n'indique dans l'amendement proposé que la création d'un crédit d'impôt ne constituerait pas une surcompensation, fragilisant le dispositif juridique de soutien à l'activité des bailleurs sociaux. Le Gouvernement a l'amendement n° 6 rectifié , nous suivons l'avis défavorable de la commission des finances, au motif que le périmètre de l'amendement est extrêmement large et conduit à supprimer toute fiscalité sur les transactions immobilières pour tous les immeubles de plus de quinze ans, quelle que soit leur fonction.

posée à la location de la résidence principale dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Nous restons cohérents avec le souci de protéger l'habitat permanent dans toutes les villes.

et les nouveaux acteurs des outils dont ils vont disposer. Certes, nous n'en sommes qu'à la première lecture au Sénat, et la route est encore longue, mais il faudra profiter de ce laps

donner l'exemple pour nos centres-villes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons une responsabilité collective dans leur fragilisation. Si nous voulons les revitaliser, nous devons donc changer complètement nos comportements. L'une des difficultés majeures de nos centres-villes et de nos centres-bourgs, c'est leur abandon par les services publics qui prend une dimension extrêmement préoccupante. Il faut arrêter cette fuite en avant ! Nous proposons quatre mesures pour les services existants. La première, c'est l'obligation d'informer les élus d'un périmètre « OSER » des projets de transfert des services publics. La deuxième obligation, c'est de justifier de l'impossibilité de maintenir le service en centre-ville. troisième obligation, c'est la possibilité pour la commune victime du transfert d'exprimer son refus, ce qui ouvre une phase de dialogue avec l'autorité responsable du service public.

Pour les services publics à venir, nous proposons d'encourager les maisons et les pôles de santé ainsi que les maisons de service public à s'installer dans les centres-villes et les centres-bourgs.

Il considère que la réaffectation de locaux vacants est bien évidemment à encourager. En revanche, on me signale que cette mesure ne relève pas de la loi. Je vous invite donc, madame la sénatrice,

Cet amendement est tout à fait bienvenu pour donner la main aux élus locaux dans ces démarches relatives au patrimoine appartenant à l'État. Président d'un département pendant sept ans, je n'ai jamais réussi à faire décroiser les propriétés départementales et de l'État

Par cet amendement, nous défendons l'idée de laisser beaucoup plus de souplesse, d'élasticité, de facilité aux élus. Si vous connaissez le visage de ces territoires malheureusement oubliés, constellés de friches, qu'elles soient agricoles, artisanales,

Le paragraphe I prévoit, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, la possibilité de demander au préfet de déroger à certaines normes qui alourdissent de façon disproportionnée la réalisation de travaux de redynamisation d'un centre-ville. Le paragraphe II exclut du champ de la dérogation plusieurs catégories de normes : les dispositions réglementaires transposant des mesures internationales ou communautaires, les normes de sécurité ou celles qui organisent les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. Nous estimons que cette exclusion n'est pas suffisante, puisqu'il pourra ainsi être dérogé aux règles d'accessibilité et aux règles environnementales, comme le confirme l'exposé des motifs. Alors que la France s'est engagée dans une démarche environnementale forte par la signature des accords de Paris, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, nous considérons que cet article envoie un bien mauvais signal. La préservation de la nature est un objectif impérieux, qui ne mérite aucune transgression, y compris au nom de la simplification et de travaux de redynamisation. Sur le fond, nous ne partageons pas l'idée que la norme est une contrainte à la libération des énergies. À nos yeux, il s'agit bien d'un outil de protection de l'intérêt général, ce qui explique qu'il est du ressort de la puissance publique de définir ces normes. Bref, la question pour nous est non non pas tellement de savoir s'il faut les supprimer ou les écarter, mais bien d'évaluer leur utilité en fonction de l'intérêt général à protéger. Sans remettre en cause le droit d'expérimentation, qui ouvre des possibilités intéressantes pour les collectivités, nous considérons que les objectifs affichés de simplification cachent en réalité une ambition

Les activités commerciales et artisanales ont besoin de souplesse et d'agilité pour assurer leur développement, en particulier dans le coeur des villes moyennes. Cependant, le champ de telles expérimentations doit être précisément défini, pour éviter que des règles impératives portant sur des domaines sensibles, comme l'hygiène ou la sécurité, ne soient levées. Je demanderai donc à la Commission de concertation du commerce de faire des propositions sur ce sujet, afin que le Gouvernement puisse revenir ensuite vers le Parlement avec une liste de domaines précis d'expérimentations possibles en la matière. En l'état, toutefois, l'article 6 et cet amendement ne peuvent être pleinement soutenus par le Gouvernement, qui en demande donc le retrait. La parole

tant ces sujets relèvent d'opinions et d'expériences locales divergentes. Je veux cependant indiquer ce qui a motivé ma position. Comme tout le monde, je crois que le patrimoine hérité doit être protégé, préservé. Ce n'est d'ailleurs pas un sujet. cours desquelles beaucoup fut détruit ou défiguré, notre pays a élaboré un cadre législatif et réglementaire protecteur, que nombre de pays nous envient et que d'autres devraient nous envier. Le Sénat a d'ailleurs récemment pris sa part en la matière. Notons cependant, pour tordre le cou à ce lieu commun sur les erreurs des élus, que ce fut souvent sur l'initiative de l'État, soucieux à une époque d'hygiène et de sécurité publique, mais aussi victime de la tyrannie de la modernité, que furent menées dans notre pays quelques hérésies destructrices au XIXsiècleet dans la première moitié du XXsiècle.

à des cadres, qui, du fait des procédures, s'inscrivent dans des calendriers qui ne sont plus en phase avec l'urgence née de la désertification des centres-villes et des centres-bourgs. Il est parfois craint que, en laissant de la liberté aux élus, des erreurs irréparables ne soient commises. Je ne le crois pas. je suis persuadé que la dévitalisation des centres est le plus grand danger à terme qui pèse sur le patrimoine. Comme je le disais hier, quand les hommes s'en vont, les pierres finissent toujours par tomber, et les meilleurs règlements n'y changeront rien. L'enjeu est donc bien de renverser cette tendance à la désertification des centres-villes et des centres-bourgs. C'est bien là le plus grand péril qui guette notre patrimoine. Et la meilleure réponse, c'est bien le retour des habitants. Il faut donc, certes, un cadre conservateur et exigeant : il existe, et personne ne souhaite sa remise en cause. Mais il faut aussi, dans la concertation et dans un esprit contractuel, laisser aux élus une capacité de discernement et d'adaptation. Bref, il faut leur faire confiance

laissés par les femmes et les hommes qui ont vécu ici, de la préhistoire à nos jours. Le patrimoine se construit au quotidien. Et il se préserve sans relâche contre les agressions. » C'est par ces mots que M. Martin Malvy, président de Sites et Cités remarquables de France, a son rapport remis au ministère chargé des affaires étrangères et consacré au rôle des patrimoines dans l'attractivité touristique de notre pays. Il est vrai que les règles en matière de protection patrimoniale peuvent paraître exigeantes. Mais c'est aussi grâce à ces règles que, au cours des décennies qui viennent de s'écouler, nous avons pu sauver un patrimoine inestimable pour nos villes, pour certains de nos villages et pour nos petites cités de caractère.

comme de nombreux savoir-faire qui en dépendent. Aussi, capitaliser sur les atouts culturels architecturaux et historiques des centres-villes représente, certes, un investissement initial, mais se révèle par la suite très positif,

structurantes proposées par ce texte et qu'il est urgent de mettre en place. Je le constate dans mon département de la Drôme, où trois villes ont d'ailleurs été retenues dans le cadre du plan Action coeur de ville : Valence, Romans, Montélimar. est tout aussi crucial d'agir pour les petites villes et les bourgs ruraux. Ceux-ci connaissent à leur échelle des difficultés comparables et souhaitent redonner vie à leur centre-ville ou centre-bourg délaissé, mais qui a souvent un cachet historique, quand ce n'est pas une valeur patrimoniale reconnue. C'est pour cela que j'interviens plus spécifiquement sur l'article 7, qui prévoit des mesures applicables au patrimoine protégé dans les zones OSER. Il a été le principal point d'achoppement de cette proposition de loi. Avant son passage en commission, nous nous sommes inquiétés des conséquences de cet article sur la protection du patrimoine dans nos territoires et sur le risque de revenir sur les dispositions équilibrées votées voilà deux ans dans le cadre de la loi relative à la liberté Nous estimions notamment que la remise en cause de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, l'ABF, initialement prévue par cet article, ou encore la mise en place de dérogations aux dispositions s'appliquant aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables n'étaient pas envisageables. Je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant que le rapporteur pour avis de la commission de la culture, Jean-Pierre Leleux, partage les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs que nous, à savoir préserver un dialogue entre toutes les parties en amont de la procédure « OSER » et lors de toutes les phases de sa mise en oeuvre : délibération et travaux.

semble à présent plus équilibrée. Elle permettra de procéder aux aménagements nécessaires pour revitaliser et restaurer les communes dans les périmètres OSER, tout en assurant la protection du patrimoine, lorsque celle-ci sera justifiée, dans les conditions prévues par la loi LCAP de 2016 : avis conforme de l'ABF, dans le cadre d'un dialogue avec les élus. Cependant, mes chers collègues, nous vous proposerons trois amendements. Le premier, que je présenterai dans un instant, vise à apporter une précision, et les deux autres tendent à garantir pleinement l'avis conforme de l'ABF. Ces amendements étant équilibrés et constructifs, nous espérons un avis favorable du Gouvernement et de la

eh bien, nous nous sommes mis d'accord et nous avons bien sûr accepté cet article 7, tel qu'il est aujourd'hui rédigé. Pour nous, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France est essentiel.

Finalement, cet article 7 de la proposition de loi nous donne l'occasion de dire que, parmi les dimensions de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, figure justement la protection patrimoniale. Nous savons bien qu'elle en est même un élément constitutif. élément constitutif. C'est un enjeu de qualité de vie, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu d'attractivité, c'est un enjeu de rayonnement. Autant de vertus que,

de la commission de la culture, et surtout sa capacité pédagogique à expliquer la complexité des dossiers patrimoniaux. Nous l'avons tous rappelé, la désertification des centres-villes a des causes économiques fortes. Le commerce de détail a été mis en péril par la multiplication des grandes surfaces, la grande distribution ayant trouvé d'énormes facilités dans les périphéries. Résultat, nos entrées de villes sont des désastres urbanistiques, où les grandes enseignes se mêlent aux affiches et aux parcs de stationnement, dans un désordre général qui va de Dunkerque à Nice. Quand on voyage en France, on a le sentiment d'entrer toujours dans les mêmes villes. Mes chers collègues, ayons l'honnêteté de dire que

termes : « Il s'agit de concilier deux impératifs qui peuvent paraître opposés : conserver notre patrimoine architectural et historique et améliorer les conditions de vie et de travail des Français. »

! Je revendique que nous ne soyons pas obligés de découvrir le paysage urbain, la citadelle et la cathédrale au milieu d'un bric-à-brac de cubes, de parallélépipèdes et de pancartes en tous genres

Ce premier amendement vise à allonger d'un à deux mois le délai dont disposera l'ABF pour porter à la connaissance des élus les documents d'urbanisme et les servitudes en vigueur existant sur la zone concernée, lors de la phase pendant laquelle la mise en oeuvre de l'OSER sera envisagée, sans être encore entérinée.

de décisions parfois épars. Un délai d'un mois risque donc d'être insuffisant. Cet allongement de délai nous semble d'autant plus utile que les ABF sont en nombre très insuffisant

Ainsi, ils doivent souvent faire appel à des vacataires n'ayant pas encore leur diplôme d'architecte. Avec la création des OSER, leur charge de travail va se trouver encore augmentée, et ils vont devoir faire face à de nouvelles obligations. Les situations de blocage ne sont pas uniquement dues, comme je puis l'entendre dire parfois, à tel ou tel trait de caractère qui serait commun à l'ensemble des ABF ; elle résulte du fait que l'on ne leur donne pas les moyens d'effectuer dans des conditions décentes leur mission. Si l'on veut favoriser un réel dialogue avec les élus, qui évitera de nombreuses situations de blocage, il me semble donc préférable de prévoir un délai convenable pour porter à la connaissance des élus les servitudes et autres documents d'urbanisme, et ainsi favoriser les discussions. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à porter à deux mois le délai dont disposera l'ABF pour porter à la connaissance des élus ces documents.

est la réalité de la situation dans les DRAC. Le Gouvernement doit satisfaire ses obligations de service public, pour permettre aux ABF de faire leur travail, en relation avec les élus. C'est absolument essentiel

Il a uniquement pour objet d'apporter une précision concernant les documents ou servitudes qui devront être portés à la connaissance des élus lors de la phase préparatoire de l'OSER, en cas d'existence de patrimoine protégé sur la zone envisagée, soit au titre des abords, soit au titre d'un site patrimonial remarquable, pour la mise en oeuvre pour la mise en oeuvre de l'opération. M. le rapporteur nous a expliqué qu'il s'agissait juste de reprendre les documents existants. Il me semble néanmoins que le texte laisse subsister une ambiguïté. En effet, il prévoit que l'ABF « dispose d'un délai d'un mois pour porter à la connaissance du maire ou du président de l'EPCI les servitudes d'utilité publique et les dispositions des documents d'urbanisme instituées dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine sur ledit périmètre ». Un doute subsiste quant au fait qu'il s'agisse des documents et servitudes existant

la saisine » de l'ABF. J'espère que cette volonté de clarification rédactionnelle ne posera pas de problèmes au sein cet hémicycle. Quel est l'avis de la commission ?

actuel de l'article 7 ne précise de quelle façon les servitudes patrimoniales seront protégées lorsque des travaux seront engagés dans le cadre d'une Le patrimoine est un élément structurant pour les centres anciens et un facteur non négligeable de retombées touristiques et économiques. Assurons-nous donc de le maintenir en état de protection optimale grâce à l'avis conforme de l'ABF, tel qu'il est prévu dans le droit commun du patrimoine. Quel est l'avis de la commission ?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

Cet amendement vise la mise en place d'opérations de revalorisation touristique en cas de refus de mise en oeuvre d'une opération de revitalisation OSER au titre de l'avis des architectes de bâtiments de France. S'il est tout à fait compréhensible que le site comprenne des immeubles ou ensembles d'immeubles protégés au titre des abords ou des sites patrimoniaux remarquables et ne puisse pas, en conséquence, être réaménagé au titre de la préservation de ce patrimoine, il faut qu'une solution puisse être envisagée pour accompagner la redynamisation de la commune. Dans cet esprit, grâce à cet amendement, une concertation entre l'architecte, la commune et le représentant de l'État dans le département accoucherait d'une proposition d'opération de revalorisation touristique pour la zone concernée, afin d'y conserver l'emploi local et d'y drainer de nouveaux flux. Le patrimoine doit être pleinement considéré comme une ressource pour les territoires- c'est parfois la seule dans les zones rurales -, dans une perspective d'aménagement et de développement socio-économique et touristique. Ces opérations globales de revalorisation touristique concernent des sites ou édifices majeurs, mais aussi des entités patrimoniales plus modestes, reconnues de préférence par un label patrimonial, qui présentent un intérêt tout particulier par leur forte singularité historique ou architecturale, dans une optique d'aménagement maillant le territoire. De tels sites ou monuments, à l'attractivité touristique potentielle ou avérée, peuvent contribuer au développement économique local s'ils sont suffisamment mis en valeur et accessibles au public. Ils doivent correspondre à des programmes d'investissement, à la fois matériels et immatériels, comprenant nécessairement plusieurs volets. Quel ? L'avis de la commission est défavorable, pour plusieurs raisons. D'abord, l'amendement manque de précision. Ensuite, on a déjà intégré un certain nombre de choses, dont l'attractivité touristique, dans les opérations de revitalisation.

est l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Il nous semble que, lorsque c'est justifié, rien n'empêche le représentant de l'État, le préfet,

Celle-ci participe à l'accès de nos concitoyens à la lecture et au savoir, mais c'est également un lieu d'animation culturelle et sociale. Au moment de

Je vous propose donc de permettre aux communes et aux communautés de communes de les subventionner- ce serait facultatif -à hauteur de 30 % du chiffre d'affaires.

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement est très attaché au soutien des librairies indépendantes. Toutefois, celles-ci, en particulier les librairies indépendantes de référence, peuvent déjà bénéficier d'une exonération de contribution économique territoriale et d'appuis des collectivités locales, dans la limite de leurs attributions, fixées au code général des collectivités territoriales, dans le cadre communautaire, qui prévoit des règles spécifiques pour la distribution d'oeuvres littéraires.

des petites villes et des centres. J'ajoute que, parfois, elles servent aussi de dépôt pour la presse. Nous sommes en train de travailler sur la crise de la distribution de la presse et, là où il y a des librairies, il y a du potentiel de diffusion de

que développent de nombreuses activités, et être dans la course et sur les marchés, avec la performance permettant d'être compétitif. L'idée proposée au de leur accorder un crédit d'impôt sur les investissements qu'ils pourraient faire pour, justement, être sur le marché numérique. Ce crédit d'impôt avait été initialement envisagé à hauteur de 50

sensible au reproche qui lui a été fait, la commission des finances a émis un avis de sagesse. Quel est l'avis du Gouvernement ? Vous ne serez

Vous ne serez pas non plus surpris si j'ajoute que le Gouvernement n'est pas favorable à la création de nouvelles niches fiscales, lorsqu'elles sont non chiffrées- j'ai néanmoins entendu quelques évaluations, qui restent d'un montant significatif -et non bornées dans le temps. Pour mémoire, toute création ou extension de dépense fiscale doit être d'une durée maximale de quatre ans, conformément à ce qui a été inscrit dans la loi Toutefois, le Gouvernement est extrêmement sensible au sujet de l'adaptation des TPE et PME, en particulier dans le domaine du commerce et de l'artisanat, au monde du numérique et à la transformation numérique.

ce n'est pas raisonnable. D'abord, la somme en question est très importante. En outre, les dépenses éligibles sont, honnêtement, très floues ; qu'est-ce que cela veut dire, pour un commerçant, d'avoir une plateforme de vente en ligne ? Cela peut vouloir désigner des choses très compliquées et coûteuses, ou des choses qui le sont beaucoup moins

avec les cadeaux qui sont faits par les différents gouvernements depuis des années aux grandes surfaces ; vous

les petits commerces indépendants, dans la ruralité ou dans les villes, ont de grandes difficultés, et, s'ils n'ont pas les moyens de faire des choses, ils disparaîtront complètement. On parle de 10 vote. Je serai toujours celle qui vous fait atterrir dans nos pays, mais je sais que c'est pour votre plus grand bonheur, tellement ils sont beaux et attirants ... Lorsque l'on achète, en France, un ordinateur de capacité correcte entre 800 euros et 1 000 euros, il vaut le double chez nous,

simplement rappeler qu'il s'agit là d'un plafond de dépense, qui permet à chaque commerçant ou artisan de définir ce qui correspond pour lui au meilleur moyen de développer son activité

à des artisans et des commerçants d'avoir l'audace de l'équipement leur donnant un temps d'avance sur d'autres concurrents. La

traitant le problème de l'outre-mer. Je suis sensible à cet argument, je voulais le dire. Je ne voterai évidemment pas cet amendement mais, plus tard, on regardera

le fait d'exonérer de cotisation foncière des entreprises est un élément qui permettrait de consolider le début d'activité. Toutefois, en l'état du texte, nous attirons l'attention sur la définition du périmètre «

une micro-entreprise sera concernée par cette exonération de CFE, et une autre ne le sera pas. Cela risque évidemment de poser, d'une part, des problèmes relationnels avec les micro-entrepreneurs concernés et surtout, d'autre part, une difficulté constitutionnelle.

Cette exonération sera effective en 2019. Dans le cas général, pour les micro-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires excéderait ce montant, un barème a été mis en place en 2014, qui vise justement à faire entrer les micro-entrepreneurs dans des conditions de lissage et d'égalité avec les très petites entreprises artisanales. Cela constitue une mesure d'équité.